Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre

l'amendement n° 104. La proposition de loi que nous examinons vise à améliorer notre système de santé par la confiance et la simplification. Nous proposons, dans le cadre de cet objectif, une avancée concrète, ouvrant un progrès et une simplification dans l'accès aux soins des usagers, qui consiste à s'appuyer sur les compétences des 100 000 professionnels de santé que sont les masseurs-kinésithérapeutes. et Territoires propose, avec cet amendement, de permettre aux patients d'accéder directement aux traitements de kinésithérapie. En effet, les masseurs-kinésithérapeutes bénéficient d'une large autonomie dans le diagnostic et dans les soins apportés aux patients, mais leur pratique est toujours soumise à prescription médicale. Cette restriction est parfois non pertinente. Elle souffre ailleurs d'exceptions dès à présent dans les cas d'urgence et dans le cadre de protocoles de coopération, pour la torsion de la cheville et la douleur lombaire par exemple. Ces exceptions sont justifiées, mais peu lisibles pour le patient. L'accès direct simplifierait et raccourcirait le parcours de soins du patient. Il permettrait aussi de pallier le risque de renoncement aux soins ou de surcoût pour le patient dans les territoires où il est difficile d'avoir accès à un médecin généraliste, bien que ce ne soit pas l'argument l'argument premier. Cette mesure ne représenterait pas de surcoût pour la sécurité sociale. Elle permettrait même des économies, même si, là non plus, ce n'est pas le but premier. Les soins concernés répondront aux référentiels émis par l'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé, comme c'est déjà le cas pour les dix séances prévues Par ailleurs, le lien avec le médecin ne serait pas rompu, puisque la prescription médicale resterait possible et le risque de perte d'informations serait évité en conditionnant le remboursement au versement du bilan et du compte rendu au dossier médical partagé et à la transmission au médecin traitant. proposons a été travaillée avec le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et les syndicats représentatifs de la profession. La parole

tel qu'il a été rédigé par la commission, vise déjà à rendre effective la faculté ouverte à ces professionnels d'adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie datant de moins d'un an. dans un objectif de pertinence des soins, qu'il était utile que le médecin traitant reste un pivot de la prise en charge des patients et permette de réguler l'accès aux soins de masso-kinésithérapie en dehors des situations d'urgence, dans lesquelles un masseur-kinésithérapeute peut déjà apporter les premiers actes de soins. La commission sollicite donc le retrait de ces amendements.

cet amendement a pour objet d'élargir la compétence des infirmiers, ainsi que des médecins généralistes, à la délivrance des autotests VIH, afin d'en multiplier les points d'accès. Comme la Cour l'a rappelé, malgré les récents progrès, la politique de dépistage connaît encore en France un trop grand retard. 170 000 personnes vivent avec le VIH dans notre pays et 6 500 découvrent leur séropositivité chaque année, on estime à 30 000 le nombre de personnes qui sont porteuses sans le savoir. C'est beaucoup trop. Pis, environ un tiers des découvertes sont trop tardives Afin d'enrayer cette dynamique, la France avait permis la vente des autotests en pharmacie. Plus de 90 000 autotests ont ainsi été vendus en 2017, mais ce chiffre est encore insuffisant. Il faut l'augmenter significativement pour améliorer le dépistage. C'est pourquoi il convient de multiplier les possibilités d'obtenir des autotests. En particulier, il nous semble pertinent d'ouvrir cette possibilité aux infirmiers et médecins, les consultations avec ces professionnels de santé offrant souvent au patient l'occasion de se confier.

de la commission ? Le code de la santé publique autorise la délivrance des autotests VIH en dehors des pharmacies, par des centres de dépistage, d'accompagnement ou de prévention en addictologie, ainsi que par les organismes de prévention sanitaire habilités. La délivrance par des infirmiers et médecins pourrait encore faciliter l'accès à ces dispositifs médicaux.

Le traitement post-exposition, ou TPE, au VIH et la prophylaxie pré-exposition, la PrEP, devaient permettre de poser un nouveau jalon dans la lutte contre le VIH, tout en améliorant grandement la vie de nombreuses personnes. Pourtant, alors que son autorisation de mise sur le marché, ou AMM, ne date que de 2016, et que l'on aurait donc pu penser que la phase de montée en puissance était encore en cours, on a noté une baisse de 27 345 prescriptions de PrEP entre 2019 et 2020. C'est beaucoup trop. n'est pas imputable aux personnes concernées. La crise de la covid a rendu manifestes à la fois l'insuffisance et la méconnaissance des possibilités d'accès à ces traitements. S'agissant tout d'abord de l'insuffisance, l'AMM européenne de 2016 prévoyait que la PrEP soit prescrite par des médecins expérimentés,

Le Portugal a pourtant trouvé une parade rédactionnelle dont nous pourrions nous inspirer. J'espère que cette question sera résolue rapidement, mais, pour l'heure, je me permets de rappeler, exemples à l'appui, que la prescription et la délivrance hors AMM restent techniquement possibles. possibles. Quant à la méconnaissance des possibilités d'accès à ces traitements, elle renvoie directement au reproche que j'ai formulé concernant le manque de stabilité et de cohérence de la politique de la France en matière d'exercice coordonné. La meilleure connaissance, en particulier des Cegidd, permettrait de remédier au moins partiellement à ce problème. Enfin, l'objet de cet amendement est de promouvoir une politique visant à multiplier les possibilités d'accès à la PrEP, ainsi qu'aux TPE. Nous sommes conscients des contraintes techniques et juridiques, notamment de droit européen, qui pèsent sur celles-ci, mais il n'est pas acceptable que la politique de lutte contre le VIH en soit compromise. Il est donc nécessaire d'autoriser rapidement cette prescription. Quel

la santé a préparé un texte réglementaire pour autoriser la prescription de la PrEP par les médecins de ville, c'est bien qu'il partage cet objectif ! Personne ne souhaitait

La profession d'infirmier sera amenée à jouer un rôle central dans la transformation de l'organisation de notre système de soins, mais aussi au regard de l'enjeu de santé publique considérable que représente la révolution démographique en cours. Dans le cadre du premier recours, de la collaboration avec le médecin traitant pour la prise en charge des patients âgés et chroniques et de leur rôle en santé publique, les infirmiers doivent voir leur mission évoluer. Alors que le programme Santé 21 de l'OMS pour l'Europe consacre le principe d'infirmier de famille ou d'infirmière référente, l'infirmier apparaît toujours, en France, comme le chaînon manquant du panorama de l'organisation des soins, alors qu'il pourrait constituer un triptyque fructueux avec le médecin traitant, d'une part, et le pharmacien référent, d'autre part, ce dernier ayant été consacré, je le rappelle, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Cet amendement vise à rattraper le retard que nous avons pris par rapport à bon nombre de nos voisins européens, en permettant qu'un patient en perte d'autonomie ou en affection de longue durée, en ALD, puisse désigner une infirmière ou un infirmier référent, afin d'assurer la coordination clinique de proximité. Il s'agit d'un mouvement tout aussi nécessaire que le développement des pratiques avancées. Madame la ministre, nous espérons que vous réserverez à cet amendement un meilleur accueil que votre prédécesseure.

Une infirmière ou un infirmier référent a toute sa place dans une CPTS, précisément pour coordonner le parcours de soins avec les autres professionnels ! Cette mesure permettrait

de loi Ma santé 2022. Comme pour la sage-femme référente, cette mesure semble répondre à un objectif louable de coordination des soins autour du patient, mais, ainsi que je l'ai dit en commission, je vois mal quelle en serait la plus-value concrète.

dont le suivi leur a été confié par un médecin. Ils réalisent le bilan, le suivi, les actions de coordination, l'éducation thérapeutique, etc. Le rôle de coordination de l'infirmier et son importance dans la prise en charge des patients sont reconnus dans les faits.

Pour travailler depuis de nombreuses années sur l'accès aux soins des personnes handicapées et sur l'évolution de la prise en charge des aides techniques, je puis témoigner qu'il est souvent très difficile pour les personnes handicapées d'obtenir des prescriptions dans des délais raisonnables.

charge par la sécurité sociale. À la suite des recommandations du rapport Denormandie-Chevalier, le ministre a lancé, en décembre 2020, un appel à manifestation d'intérêt pour l'élaboration de ce protocole de coopération sur la prescription aux ergothérapeutes. La délégation par les médecins de la prescription d'aides techniques aux ergothérapeutes sera promue dans ce cadre. À ce stade, je suis tenue d'émettre un avis défavorable, mais c'est une mesure tout à fait intéressante.

En effet, l'accès direct à l'orthophonie simplifierait et raccourcirait les parcours de soin du patient. Il apporterait également une réponse au risque de défaut de prise en charge pour les patients vivant dans des territoires où il est difficile d'avoir accès à un médecin généraliste,

Ce sont donc bien les orthophonistes qui déterminent, en autonomie, la mise en oeuvre d'un traitement, le nombre de séances nécessaires à l'issue du bilan et du diagnostic orthophonique qu'ils ont posé ou encore l'arrêt ou la poursuite des soins. Par ailleurs, le lien avec le médecin ne serait pas rompu, puisque la prescription médicale resterait possible et le risque de perte d'informations serait évité en conditionnant le remboursement au versement du bilan et du compte rendu des soins au dossier médical partagé

La commission ne voit pas d'opposition de principe à cette évolution.

y a beaucoup de médecins dans l'hémicycle et je ne veux vexer personne. Il ne s'agit pas du tout d'un jugement de valeur, mais tout

présenter l'amendement n° 20 rectifié . Aujourd'hui, l'ensemble des pharmaciens d'officines peut vacciner contre la grippe. Cette mesure a été mise en oeuvre avec succès. Afin d'augmenter la couverture vaccinale, les pharmaciens des pharmacies à usage intérieur, pourraient, eux aussi, bénéficier de cette possibilité de vacciner les patients et résidents présents dans des établissements de soins et médico-sociaux. Ce dispositif faciliterait grandement la couverture vaccinale des professionnels de santé en exercice dans les établissements de soins. Une telle évolution serait d'autant plus intéressante dans la perspective d'une vaccination de masse

du Gouvernement ? Depuis octobre 2019, la vaccination en ville est assurée par plusieurs professionnels de santé : infirmiers, pharmaciens d'officine, médecins généralistes, sages-femmes ... Il ne nous paraît pas nécessaire d'élargir la vaccination à d'autres acteurs.

à Mme Émilienne Poumirol. Cet amendement vise à supprimer l'article 3 de la présente proposition de loi, qui concerne la procédure de recrutement des praticiens hospitaliers,

je ne puis que me montrer sensible aux arguments qui le sous-tendent et qui évoquent toute la difficulté du Parlement à se prononcer sur une législation en morceaux, discutée tantôt dans une proposition de loi, tantôt dans des ordonnances en cours de rédaction.

la gestion des ressources humaines médicales. Il tend également à clarifier le rôle de l'établissement support et des établissements parties, pour accompagner efficacement de nouvelles organisations territoriales et le soutien à la construction progressive des filières de soins, telles qu'elles sont définies dans le projet médical partagé. cet amendement imposent au groupement non seulement de définir une politique territoriale de gestion des ressources humaines médicales, afin de définir les modalités les plus à même de répondre à ces enjeux, mais aussi d'établir des règles de fonctionnement qui puissent s'appliquer à chacun. L'implication de la commission médicale de groupement est essentielle pour garantir sa cohérence avec la stratégie médicale.

de l'offre territoriale de santé nous semble indispensable à la réussite du parcours de soins, ainsi qu'à la meilleure allocation des deniers publics. Mais, contrairement à la Cour ou au Gouvernement, nous ne sommes pas favorables, à ce stade, à des dispositions qui atténuent la volonté des établissements parties au profit des établissements supports. La dérive léonine des GHT vient d'une lacune dommageable de la loi Touraine, qui n'avait pas cru bon de les doter de la personnalité morale. En l'absence de cette dernière, que rapporteur du texte à l'époque, les groupements ne peuvent que fournir le prétexte à la captation de l'activité par les structures de taille importante, au détriment des établissements de proximité.

Poncet Monge. L'article 4, animé par la volonté de centraliser au sein de l'établissement support du GHT les décisions de créations de postes de praticiens hospitaliers des autres établissements parties, a été fortement contesté par les professionnels de santé et par certaines fédérations. Tout comme l'article 7, qui prévoyait l'intégration forcée par des directions communes, cet article devrait être supprimé. De façon plus générale, toute modification des prérogatives ou obligations des GHT nous apparaît prématurée au regard du faible recul et de la forte hétérogénéité des groupements, dont certains sont faiblement efficients ou présentent

marche sur le terrain, contre la volonté des acteurs de proximité et leur analyse des besoins de santé de territoires moins gigantesques. Force est aussi de reconnaître qu'aucun dispositif ne saurait être vertueux sur fond d'insuffisance chronique de financements. La perte d'autonomie des petits établissements de santé, qui ne tiraient guère de bénéfice du groupement, notamment en termes de mutualisation du personnel en cas de pénurie, s'est souvent accompagnée de fermetures préjudiciables aux territoires. Le niveau de déconnexion du terrain était prévisible quand un seul GHT couvre l'ensemble d'un territoire vaste comme l'ancienne région d'Auvergne

de sortir d'une conception exclusivement descendante des schémas de santé- de l'ARS vers les établissements -, en permettant justement que les diagnostics territoriaux, qui sont aujourd'hui inégalement réalisés, contraignent l'ARS dans son pilotage. Pour ces raisons, la commission demande le

Lors de la crise sanitaire, plus de 16 000 volontaires non soignants ont proposé leur aide auprès de l'AP-HP. Cet élan de solidarité est honorable, et nous devons le soutenir. Les dispositions de cet amendement ne vont en aucun cas à l'encontre des centaines d'associations présentes dans les établissements de santé.

L'action bénévole n'est pas réglementée non plus dans les Ehpad, où la création d'une convention de partenariat ou d'une charte définit les modalités de l'intervention des bénévoles. Au sein des établissements de santé, les associations organisent l'intervention des bénévoles. Les nombreux volontaires non soignants, s'ils ne sont pas inscrits dans des associations, sont donc en dehors du cadre légal. Ainsi, le rejet du bénévolat individuel semble aller à l'encontre de la situation actuelle dans les centres de santé et dans les Ehpad. Afin de prendre en considération l'agilité souhaitée par les bénévoles individuels, sans pour autant empêcher dans sa totalité leur intervention dans les établissements de santé, notre amendement vise à rétablir l'article 4 , avec des ajouts inspirés de l'encadrement existant dans l'article L. 1110-11 du code de la santé publique. Lors de l'examen du texte en commission, la suppression de cet article a été motivée par le besoin de formation des bénévoles. dispositions de notre amendement y répondent. Nous souhaitons que le bénévolat individuel puisse être réalisé dans les établissements de santé, en complémentarité avec les associations, et dans le respect des missions de chacun. en ajoutant une obligation de formation par les associations et les établissements de santé eux-mêmes, en s'assurant de la non-interférence avec la pratique des soins médicaux ou paramédicaux et de l'encadrement par un référent, nous pensons que le bénévolat individuel pourra être un soutien important pour les associations et les établissements de santé.

Madame Cohen,

Si nous saluons bien sûr l'élan solidaire fort qui a permis à des soignants de venir prêter main-forte dans les établissements de santé en cette période de crise, nous nous opposons à l'institutionnalisation d'un statut de « médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole ». Pérenniser ce statut revient à considérer le bénévolat comme un supplétif aux carences en ressources humaines constatées depuis de longues années. Ce n'est pas autre chose que du salariat déguisé. De plus, la proposition de loi ne prévoit pas les conditions de leur intégration au sein des équipes médicales et du projet médical d'établissement. Elle ne précise pas non plus les conditions d'engagements ni les modalités d'encadrement de ces bénévoles.

pareil ! Nous avions salué l'initiative de la commission, qui visait à permettre l'intervention des bénévoles dans les établissements de santé.

bénévoles dans les établissements de santé, y compris pour des missions relevant du service public hospitalier, et non pas seulement dans le cadre des activités dévolues aux associations de bénévoles. telle pratique, qui est marginale, nous le savons, ne constitue en rien une réponse adéquate ou même, comme vous le supposez, un simple palliatif au problème de la démographie médicale à l'hôpital. Il serait d'ailleurs souhaitable que ces interventions soient ciblées sur des missions complémentaires et ne

de « participer à l'exercice des missions générales de ces établissements et de celles attachées au service public hospitalier. » Il est tout de même difficile de faire plus large ! Un deuxième problème est lié aux raisons qui sous-tendent cette mesure. À cet égard, permettez-moi de citer les auteurs de l'amendement adopté à l'Assemblée nationale de contribuer au « renforcement des ressources médicales des établissements publics de santé dans l'intérêt du service public hospitalier et dans le contexte actuel de la démographie médicale

C'est pourquoi, à défaut d'une suppression de cet article, cet amendement vise à instaurer un garde-fou basique, pourtant essentiel : il s'agit d'empêcher que les contrats conclus avec les praticiens exerçant à titre bénévole ne se substituent aux postes d'agents titulaires laissés vacants.

assurer des missions de soutien et d'animation et celle des professionnels de santé qui viennent assurer des missions de soins en complémentarité des équipes en place. Dans les deux cas, ces interventions sont encadrées par des conventions avec l'établissement concerné. Contrairement à ce que vous affirmez, il s'agit non pas de pallier une pénurie de moyens, mais de répondre à une volonté d'engagement citoyen,

L. 6152-5-1 du code de la santé publique et adoptées dans le cadre de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. En effet, l'application de cette loi devient urgente pour éviter le départ massif de professionnels des hôpitaux publics, en particulier pour les établissements situés dans ou à proximité immédiate d'une zone de revitalisation rurale, une ZRR, comme le centre hospitalier Émile-Roux du Puy-en-Velay. Les forts avantages fiscaux de la ZRR créent alors une réelle distorsion de concurrence, au détriment des établissements publics de santé, dont les praticiens sont parfois activement démarchés par des cabinets de conseil. Cet amendement tend à accorder un ultime délai au Gouvernement pour prendre enfin les mesures d'application de ces dispositions, pendant le premier semestre de 2021. Quel

et l'activité libérale exercée par un praticien salarié d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un Espic. L'exercice de l'activité libérale est plus aisé pour le praticien lorsque celui-ci exerce en hôpital public. Cet amendement Cet amendement vise à corriger cet écueil, en recentrant l'activité hospitalière de ces praticiens sur le strict service public hospitalier et en permettant aux praticiens salariés d'un Espic de pratiquer des dépassements d'honoraires, dans la limite des dispositifs de maîtrise prévus par la convention médicale.

À la différence des praticiens du secteur public hospitalier, les praticiens des Espic ne peuvent avoir d'activité libérale. Il existe donc une inégalité de traitement dans la loi entre l'activité libérale exercée par un praticien hospitalier d'un établissement public de santé et l'activité libérale exercée par un praticien dans un établissement de santé privé d'intérêt collectif. Je vous le rappelle, les Espic jouent un rôle essentiel au côté des hôpitaux publics et des cliniques privées. Le présent amendement vise donc à faire évoluer cette situation paradoxale, pour permettre aux praticiens des Espic d'exercer une activité libérale avec dépassement d'honoraires, en marge de leurs activités de service public hospitalier, dans le cadre de leur exercice en Espic, avec, pour contrepartie, un reste à charge financier nul pour les patients. Une égalité de traitement doit être rétablie. Je le rappelle, les Espic représentent 8 % de l'offre de soins et sont le plus souvent créés par des fondations reconnues d'utilité publique. Ils sont souvent à la pointe de la technologie et de l'innovation.

il tend à renforcer l'attractivité des métiers, en permettant aux médecins qui travaillent en Espic ou en établissement public d'accéder à une égalité de traitement absolument nécessaire.

parole est à Mme Michelle Meunier, sur l'article. Nous ouvrons le chapitre consacré à la gouvernance des établissements publics de santé, dans cette proposition de loi qui se veut être la traduction sur le plan de l'organisation des soins des conclusions du Ségur de la santé. Dans l'esprit des soignants comme dans celui de bon nombre de nos concitoyens, attachés au bon fonctionnement du système de santé, le Ségur s'est soldé par une revalorisation. chez nombre d'agents du secteur social et médico-social, le sentiment d'être des oubliés du Ségur perdure. Ce ne sont pas seulement des oubliés, ce sont aussi des déçus. sont déçus par une disparité de traitement qui ne connaît pas de justification et entraîne une profonde désorganisation du médico-social. Sur le terrain, les conséquences sont désastreuses et source d'incompréhension pour ces soignants non médicaux, qui portent aussi blouse blanche et qui interviennent non pas en établissement hospitalier, mais dans des centres de soins, des foyers d'accueil médicalisés, des maisons d'accueil spécialisées ou encore dans des services de soins infirmiers à domicile. Selon qu'elles exercent- en effet, ce sont principalement des femmes -leur métier dans ces structures plutôt qu'à l'hôpital, elles ne bénéficient pas de la revalorisation salariale. C'est le cas notamment l'établissement de Saint-Brévin-les-Pins, dans mon département de la Loire-Atlantique, dont les agents brûleront symboliquement leur diplôme demain devant la sous-préfecture de Saint-Nazaire. Le geste est fort. Pour toutes celles et tous ceux qui agissent au quotidien pour un accès aux soins de qualité auprès des personnes âgées et/ou en situation de handicap, on enfonce un peu plus le clou de la dévalorisation de leur métier, dont la pénibilité est avérée. Pour les associations qui les emploient, parfois déjà fragilisées par les surcoûts de la crise, il y aura, à plus ou moins long terme, des répercussions sur le recrutement, mais aussi sur la fidélisation des professionnels,

Quel est l'avis de la commission ? Le Gouvernement inaugure par cet amendement une série de propositions relatives à la gouvernance hospitalière, qui visent tout simplement à ne pas tenir compte des travaux de notre commission. Les amendements de rétablissement, s'ils relèvent d'une position parfaitement acceptable en soi, peuvent révéler la précipitation, voire la paresse, de leurs auteurs, lorsque l'argumentaire n'a manifestement pas tenu compte des ajouts opérés par la commission. En l'occurrence, les modifications apportées à l'article 5 avaient justement pour objet de renforcer le rôle du chef de service, en précisant son positionnement par rapport au chef de pôle, ce que la rédaction initiale négligeait de faire. Par ailleurs, elles matérialisent une recommandation forte du rapport Claris, en approfondissant la délégation de tâches vers les chefs de pôle, qui disposeront ainsi d'une enveloppe leur permettant d'engager des décisions financières dans un montant fixé par arrêté. La commission est donc défavorable à cet amendement du Gouvernement.

de santé pointaient pour les personnels, y compris médicaux, l'insuffisance d'informations sur les orientations stratégiques de l'hôpital, sur l'actualité de ces projets ou encore sur les éléments d'actualité du pôle. Ce rapport mettait de plus en avant les difficultés pour les instances représentatives du personnel, qui n'étaient que peu informées du dialogue existant au sein des pôles, notamment en ce qui concerne les actions directement menées par le chef de ce pôle. Les rencontres et les échanges avec les personnels hospitaliers ont confirmé l'ensemble de ces critiques et de ces dysfonctionnements des pôles médicaux. Le rapport et les recommandations de Mme Nicole Notat, à l'issue du Ségur de la santé, soulignaient également que la structuration des hôpitaux en pôles s'est souvent par raison, voire par contrainte. La multiplication des strates d'organisation a entraîné une déconnexion des prises de décisions avec le terrain. Par conséquent, nous proposons de tirer l'ensemble des conclusions qui s'imposent et de supprimer les pôles d'activité, afin de renforcer par ailleurs la commission médicale d'établissement, seule instance élue et démocratique de l'hôpital. L'amendement Bernard Jomier. Au terme d'un sondage organisé par la mission du professeur Claris, il apparaît que 65 % des personnels hospitaliers estiment que les services n'ont pas trouvé de voix d'expression au sein des pôles. Aussi, comme j'ai pu le dire au début de la séance, au cours de la discussion générale, l'intention des auteurs de l'article 5 est louable, puisque ce dernier réaffirme le rôle des services et du chef de service, suivant ainsi une recommandation du rapport Claris. Le service de soins doit être le niveau de référence pour les équipes soignantes comme pour les patients au sein de la gouvernance de l'établissement. Cependant, des voix s'élèvent parmi les personnels hospitaliers pour que cette réforme ne s'arrête pas au milieu du gué. Leurs craintes sont légitimes, car revaloriser, sur le papier, du rôle des services, sans modifier le rôle et le champ d'intervention des pôles d'activité, risquerait d'entraîner une forte désillusion. La consécration du pôle d'activité comme maillon matriciel de l'hôpital public, engagée au début des années 2000 et achevée en 2007, a découlé de l'exigence de l'époque de retenir un échelon intermédiaire entre le service et la direction, afin de permettre une certaine déconcentration de la gestion, tout en garantissant la liberté d'organisation de l'hôpital. On en connaît bien les écueils : verticalité de la prise de décision, approche trop managériale et gestionnaire, loin du vécu des personnels soignants, qui peinent à faire entendre leur voix. le rapport Claris est clair à ce sujet : la solution réside justement dans le travail sur la maille décisionnelle, évacuant tout débat quant à la maille organisationnelle. Le rapport de la commission précise d'ailleurs que, « de l'avis général des directions d'établissement, la pertinence du pôle d'activité comme maille organisationnelle n'a jamais été discutée part des directions d'établissement, ce n'est pas extrêmement surprenant ... Cependant, il nous semble regrettable de mener ce débat aussi rapidement. Si la solution n'est sans doute pas de procéder à la suppression des pôles- vous l'aurez compris, mes chers collègues, je présente un amendement d'appel -, il nous semble nécessaire d'avoir un véritable débat quant quant à cette maille organisationnelle. Les personnels hospitaliers ont ressenti pendant la crise de la covid que la verticalité qu'il connaissait pouvait s'estomper au profit d'un travail collectif et d'un dialogue plus horizontal. Avoir ce débat, c'est aussi les entendre. L'amendement

toute la place qui doit être la sienne du point de vue du fonctionnement médical de l'établissement- le nouvel article 5 de la proposition de loi y contribue fortement -, nous ne sommes pas défavorables au pôle d'activité comme échelon organisationnel. Je rappelle d'ailleurs aux auteurs de ces amendements, Mme Cohen et M.

opportune, en ce qu'elle alourdirait les structures de direction du service et exposerait potentiellement ce dernier à un conflit de hiérarchie entre chef de service et chef de service adjoint.

à celui que nous entendons envoyer au travers de l'article 5. Alors que nous tentons de revaloriser le chef de service, doubler sa hiérarchie fonctionnelle par la création, dans la loi, d'un poste d'adjoint au chef de pôle,

pour établir les professionnels de santé au sein de la gouvernance des établissements. C'est une mesure tout à fait positive, mais qui nous sommes largement insuffisante si elle ne s'accompagne pas d'un renforcement de la démocratie sanitaire. Nous proposons donc d'accorder aux chefs de service une légitimité démocratique qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Pour ce faire, nous proposons de substituer à leur nomination leur élection les membres de la commission médicale d'établissement. Aux termes du présent texte, les chefs de service sont nommés par le directeur de l'établissement hospitalier, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de composante ou d'unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique. Pour nous, cette nomination s'apparente davantage à une cooptation, ce que nous n'approuvons pas. Par notre amendement, nous souhaitons donc éviter l'entre soi des professionnels de santé et renforcer les pouvoirs de la commission médicale d'établissement, instance représentative de la communauté médicale, pharmaceutique et odontologique. De plus, nous proposons que, dans les centres hospitaliers universitaires, les chefs de service soient élus pour quatre ans, avec un binôme titulaire-remplaçant composé à parité d'une femme et d'un homme. Enfin, nous entendons encadrer

En revanche, il est réducteur en ce qu'il exclut le directeur de l'UFR de santé concernée lorsqu'il s'agit de nommer lesdits chefs de service en médecine, en odontologie et en pharmacie dans les centres hospitaliers et universitaires.

du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de composante ou d'unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.

comme structure interne des pôles d'activité des centres hospitaliers et universitaires, alors que, jusqu'alors, la structuration interne de prise en charge du malade au sein des pôles était laissée à la discrétion des établissements hospitaliers, dont certains avaient supprimé le terme « service », en utilisant l'appellation « unité interne », plus réductrice. 5 rétablit également, et fort justement, l'appellation « chef de service », plus valorisante et plus reconnue dans le monde hospitalier, y compris à l'international, qui avait elle aussi plus ou moins disparu dans certains centres hospitaliers. En revanche, en l'état, cet article est réducteur, puisqu'il exclut le directeur de l'UFR de santé concernée lorsqu'il s'agit de nommer lesdits chefs de service en médecine, en odontologie, en pharmacie dans les centres hospitalo-universitaires. Il est aussi peu cohérent avec le même article L. 6146-1 du code de la santé publique, dont il est la déclinaison. En effet, dans plusieurs alinéas, cet article associe systématiquement le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, que ce soit pour définir le projet médical d'établissement,

pharmaceutique et odontologique. Tel est le sens des ordonnances Debré, dont l'objectif était de renforcer les interactions entre centres hospitaliers et universités, qui définissent les missions des centres hospitaliers et universitaires. La désignation d'un chef de service universitaire aura un impact en matière de formation et de recherche. Cette désignation faite conjointement par le directeur de l'établissement, le président de la CME

Jomier. Le chef de service est un interlocuteur privilégié, au centre de l'organisation de travail. Il apporte une réelle plus-value sur le terrain des soins, compte tenu de sa connaissance des équipes et des besoins du service. Désigner un chef de service, c'est désigner un professionnel de terrain, au plus proche des équipes de soins. Il paraît inapproprié que les chefs de pôle, instances administratives et organisationnelles, puissent interférer dans la nomination des chefs de service. Le service étant l'unité la plus à même de répondre avec pertinence aux prises de décision et à la mise en oeuvre de la politique médicale, son chef doit être nommé par les personnes concernées, pour davantage de confiance et de coordination. L'amendement n° 169, présenté par M. Jomier,

Cette commission est un lieu de réflexion, de partage et une force de proposition de l'ensemble des professionnels paramédicaux de l'hôpital. Elle témoigne de leur implication dans le développement de la qualité de la prise en charge des patients à l'hôpital. Pour que la décision relative à la nomination des chefs de service soit réellement partagée,

Mme Cathy Apourceau-Poly. Dans la continuité des amendements déposés par nos collègues et en cohérence avec notre projet de refonte de la gouvernance hospitalière, visant à rétablir une véritable démocratie sanitaire, nous proposons que, en amont des nominations des chefs de service, une concertation avec les personnels du service concerné soit organisée. La proposition de loi renforce l'autorité des chefs de service dans la gouvernance des établissements publics de santé. Il s'agit d'un progrès par rapport à la gouvernance de gestionnaires éloignés de nos services. Ce système existait auparavant, et nous avions pu observer les défauts d'un tel mode de fonctionnement, avec les dérives personnelles de certains médecins et une mise en concurrence des services entre eux. C'est la raison pour laquelle nous sommes favorables au renforcement de la place des représentants du personnel dans les instances. Par cet amendement, nous proposons d'inclure une concertation avec les personnels

L'article 5 répond à une attente des personnels hospitaliers, en réaffirmant la place de référence des services et du binôme du chef de service et du cadre de santé. Nous nous en félicitons, tout comme nous nous félicitons que l'article prévoie que les chefs de service seront nommés par décision conjointe du directeur d'établissement et du président de la commission médicale d'établissement. Cette codécision constitue une première avancée, avec la concertation prévue avec les personnels affectés dans le service. Mais sa portée sur le partage de la décision est réduite par l'amendement adopté en commission, qui a pour objet que, en cas de désaccord, la décision revient à l'une des parties, en l'occurrence le directeur ou la directrice d'établissement.

amendements suivants -, qui respecte le texte de la commission, en prévoyant bien que la décision en dernier recours appartient au directeur d'établissement, en cas de désaccord entre les autorités de nomination. J'ajoute que cette précision est d'autant plus utile que ces autorités seraient désormais au nombre de trois

semble louable, mais ce changement créerait, à mon sens, une double confusion : d'une part, la partie réglementaire du code de santé publique- et la principale partie de sa partie législative -faisant mention de « centres hospitaliers universitaires », il ne me paraît pas souhaitable que deux deux dénominations coexistent pour désigner la même entité ; d'autre part, l'introduction de ce « et » semble atténuer le partenariat nécessaire qu'abrite le CHU entre pratique hospitalière et recherche médicale, ce qui me semble inopportun. La commission émet donc un avis défavorable

ne me paraît pas applicable, dans la mesure où, je le répète, le chef de service est d'abord une autorité fonctionnelle chargée d'appliquer la ligne de gouvernance de l'hôpital à l'échelle du service. Bien qu'il soit fondamental que les liens avec son équipe soient de bonne qualité, il ne me semble pas raisonnable que la loi doive s'en préoccuper en amont de sa nomination, par une concertation dont les résultats ne lieront pas les autorités de nomination. La commission émet donc un avis défavorable sur cet

ne pas les intégrer à la concertation, ce serait adresser un très mauvais signal aux jeunes internes, qui contribuent activement à l'activité médicale des services et des hôpitaux.

concertation menée au sein des services. Or cette préoccupation me paraît satisfaite : l'alinéa 9 de l'article 5 vise bien, au sein du service, l'encadrement des internes

commission ? Cet amendement tend à ériger au rang législatif l'une des missions qui incombent naturellement aux chefs de service et aux cadres de santé dans la gestion quotidienne des équipes.

totalement volontaire. L'initiative en reviendrait au chef d'établissement, s'appuyant sur les avis conformes de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Cette expérimentation aux contours très bien définis serait prévue pour une durée de trois ans et ferait l'objet d'une évaluation.

Bernard Jomier. L'enjeu de l'adaptation du système de santé, notamment de l'offre de santé hospitalière, aux besoins de santé spécifiques de la population, a été conforté par tous les grands projets de loi depuis la

la volonté du législateur est bien de tenir compte de l'évolution des données démographiques, sanitaires et sociales de la population, pour y adapter l'offre de soins. Or, dans les faits, cet objectif ne semble revêtir qu'une réalité formelle. Les communautés médicales et de soignants, en particulier à l'hôpital, ressentent ce décalage dans leur pratique quotidienne. Elles souhaitent que les besoins de santé soient davantage évalués et objectivés à l'échelle de l'établissement de santé : ce serait la première étape d'une adaptation de l'organisation et des moyens,

les besoins de santé de la population font l'objet d'un diagnostic et d'une révision réguliers, à échéance maximale de cinq ans. Ce faisant, l'on adapte les politiques régionales et locales d'offre de soins pour répondre aux besoins de la population.

recueillies entre le 1 octobre et le 31 décembre 2020, montre que presque 42 % des personnes en situation de handicap n'ont pas pu recevoir leurs soins.

différents services doivent pouvoir s'adapter aux particularités de chacun : difficultés dans l'explication des symptômes, mauvaise compréhension des signaux de mal-être, intolérance à la lumière, au bruit, etc. Bien que la loi impose la prise en compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap à chaque étape du parcours de soins, il nous semble important de préciser de nouveau par écrit, dans chaque projet d'établissement, les dispositifs à installer ou à travailler

de formation, de soins et d'innovation en santé. L'appellation « centres hospitaliers et universitaires » serait ainsi conforme à l'article L. 6142-3 du code de la santé publique et aux articles L.

Le projet médical des CHU comprend l'articulation avec les objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation, qui ne sauraient entrer en contradiction avec le contrat de l'université. Pour renforcer les interactions entre centres hospitaliers et universités, qui sont au coeur des missions des CHU, nous proposons d'associer également le président de l'université avec laquelle le centre hospitalier a passé la convention prévue à l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, pour préparer les objectifs stratégiques

La qualité de la formation dépend donc en grande partie des moyens humains et financiers dont disposent les hôpitaux. On ne peut que le déplorer : parfois, les étudiants en médecine comblent les déficits en personnel de l'hôpital.

le président de cette instance dans ses prérogatives actuelles, tant comme coordonnateur de la politique médicale de l'établissement que comme responsable, avec le directeur, de l'élaboration du projet médical.

Même avis.

une sous-commission mixte de la CME réunissant des praticiens, soignants, usagers et représentants de ville, fragilise ce

quant à la création d'une commission médico-soignante. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes appliqués à apporter, à l'article 6, les modifications requises pour que sa création et son maintien restent soumis à la volonté conjointe des deux commissions formant cet La suppression de cet article poserait un problème plus important encore. Tel qu'il est issu des travaux de la commission, il établit- enfin ! -, à la demande des personnels paramédicaux, le principe d'une élection du président de la commission des soins infirmiers ; bien entendu, il ne me paraît pas

sociales du Sénat, qui permet d'autoriser, sous la forme d'un droit d'option, le regroupement de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, pour les seuls établissements qui le souhaitent.

sont difficiles à évaluer. Or ce sont précisément ces bénéfices qui ont justifié sa mise en oeuvre, dans le cadre de la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. pour intérêt de mutualiser les ressources, quelles qu'elles soient, pour créer une dynamique de territoire autour d'un projet médical partagé, il n'a pas pour autant de personnalité morale et n'a pas à décider de l'affectation de telle ou telle ressource.

de tels procédés traduisent une confusion entre mutualisation et transfert de compétence. Les hôpitaux qui ne sont pas support perdent ainsi tout pouvoir et le conseil de surveillance n'a plus aucun regard sur les mutualisations.

une manière de centraliser les décisions et la gestion relatives aux établissements support. Or il convient de préserver leur autonomie et de conforter leur capacité à répondre aux besoins des territoires en matière de soins.

Cet amendement, qui vise à supprimer l'association de la commission des soins infirmiers à la discussion du projet médical partagé du GHT, laquelle

et vice-présidée par le coordinateur général des soins, lequel, à l'inverse du président de la CME, n'est pas élu par les membres de la commission, mais désigné par le directeur. Cela véhicule un message d'irresponsabilité vis-à-vis des soignants non-médecins qui n'est pas très valorisant. Du point de vue de la réalisation, ensuite, l'idée de fusionner les deux commissions peut sembler louable pour lutter contre les silos ; en l'espèce, elle est inutile. Le président de la conférence nationale des CME des centres hospitaliers pointe avec justesse plusieurs failles pratiques : que dire de l'effectivité d'une commission, dont le président serait élu par les membres de la CME et le vice-président désigné par le directeur d'établissement ? ? Que dire de l'effectivité d'une commission, dont le président et le vice-président n'entretiendraient pas de lien hiérarchique et conserveraient leurs compétences respectives d'anciens présidents des commissions concernées ?

et sa naissance n'est clairement pas souhaitable. Je reprends, en conclusion, les mots du président de la conférence nationale des CME des centres hospitaliers : « Tout cela, en vérité, n'a pas de sens ! » Quel

qui renforce le droit des commissions constituantes d'en sortir, dès lors que la majorité de l'une d'entre elles le souhaite. L'avis est donc défavorable.

pourtant, les projets de restructuration hospitalière sont toujours à l'ordre du jour, prévoyant la fermeture de centaines de lits et la suppression de nombreux emplois hospitaliers. J'ai à l'esprit l'exemple de l'hôpital Bichat, où ma collègue Laurence Cohen s'est rendue pour soutenir les personnels et les usagers qui refusent sa fusion

davantage, me semble-t-il, sur la pertinence de faire se croiser encore plus de malades au même endroit. Surtout, la fermeture d'hôpitaux, de services et de lits est en complète contradiction avec les besoins. Cet exemple parisien est loin d'être un cas isolé. Dans le département du Val-de-Marne, un projet de fusion de la Fondation Vallée et de l'hôpital Paul-Guiraud a été présenté aux représentants du personnel. Des projets de restructuration existent aussi en Seine-Saint-Denis, dans l'Essonne ou dans le Pas-de-Calais, où le nouvel hôpital de Lens va être construit

hospitaliers qui ont été fermés en 2019 et quatre mille en 2018. Ces chiffres sont

Sur le terrain, l'inquiétude remonte chez les soignants, les responsables d'hôpitaux et les élus locaux, qui estiment que rien n'a changé. Nous demandons donc l'instauration d'un moratoire sur l'ensemble des projets de fermeture de services, de lits et d'établissements pour lancer un débat national sur l'importance des services de santé et l'enjeu de maintenir des places pour les patientes et les patients. Quel

Il ne faut pas oublier que l'offre de soins, comme tout maillage, se doit de répondre aux évolutions démographiques, économiques et sociales des territoires qu'elle couvre.

Cet amendement vise à rétablir l'article 7 dans la rédaction adoptée par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, prévoyant la poursuite de l'intégration des GHT par le prisme des directions communes. Les postes de direction vacants d'établissements parties au GHT seront, dans un premier temps, confiés à l'établissement support pour une durée d'un an, à l'issue de laquelle le directeur de l'ARS pourra décider de poursuivre ou non la direction commune, après avis

à partir de l'établissement support, de poursuivre l'activité dans certains établissements isolés, sans avoir recours à l'intérim. À mon sens, un GHT

et le règlement intérieur qui vient la compléter. Toutefois, pour permette de concilier la nécessaire autonomie des établissements et le développement de synergies territoriales

l'interopérabilité, la réversibilité, la convergence et la sécurité des systèmes d'information en santé. Pour autant, le manque d'efficacité actuelle dans l'échange d'informations entre professionnels de santé, parfois au sein d'un même établissement, nécessite d'inscrire explicitement dans la loi la recherche d'interopérabilité. Cet amendement prévoit donc que l'établissement support des GHT s'assure que le système d'information hospitalier soit non seulement convergent, mais également interopérable. S'il était voté, cet amendement permettrait à chaque GHT d'être acteur de cette interopérabilité- elle est cruciale pour améliorer notre système et simplifier les échanges entre professionnels de santé.

de réelles difficultés subsistent ou sont apparues dans plusieurs établissements et groupements hospitaliers de territoire. Ces difficultés, relevées tant par l'inspection générale des affaires sociales dans son rapport portant bilan d'étape des GHT de décembre 2019 que par la Cour des comptes dans son rapport annuel d'octobre 2020, sont liées à des problématiques de dimensionnement, de pertinence territoriale, de management ou de cohérence avec les filières de soins. La disposition nouvelle prévue dans cet amendement vise à valoriser la la dynamique née des accords du Ségur de la santé et à rendre tangible la confiance placée dans les acteurs de santé du territoire. En outre, elle répond pleinement à l'objectif de simplification des organisations.

Fort heureusement, l'Assemblée nationale a supprimé toute la partie concernant ce numéro, lequel n'avait rien d'unique, puisqu'il s'ajoutait au 15, l'actuel numéro du SAMU, au 112, le numéro européen d'urgence, sans parler du 17, du 18, du 39 66, du 115, etc.

article 7 ! La proposition de loi a souvent été l'occasion de faire passer en catimini des mesures disparates, mal préparées et non concertées. L'article 7 en est l'exemple : introduit par un amendement en commission à l'Assemblée nationale, il entendait créer un numéro national unique santé dévolu aux services d'accès aux soins, incluant le numéro d'aide médicale d'urgence. Nous partageons la nécessité de mieux coordonner la gestion des urgences, comme celle de la permanence des soins, mais cet article n'unifie pas les urgences- cela nous semble pourtant constituer un préalable -, tout en incluant la permanence des soins, ce qui inquiète légitimement beaucoup d'acteurs, des médecins généralistes aux sapeurs-pompiers.

et en ignorant les alertes des acteurs. Sur le fond, mettre en place un numéro unique santé incluant le seul service d'aide médicale d'urgence n'apporte pas de réponse aux problèmes de coordination des urgences, qui sont connus de longue date. Nous aurions ainsi, d'un côté, un numéro unique santé pour les problèmes de santé urgents comme pour ceux qui ne relèveraient pas d'une urgence proprement dite et, d'un autre côté, d'autres numéros de recours d'urgence. Où est donc la simplification ? Comme le notait la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, créer un numéro santé 113, c'est renoncer à faire du 112, numéro d'urgence européen, le numéro unique pour tous les appels de secours d'urgence relevant des SAMU, de la police, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers,

la rédaction finalement adoptée par l'Assemblée nationale ne fait plus référence à un numéro unique pour laisser de la souplesse en fonction des organisations territoriales préexistantes.

Mais nous ne pouvons pas nier non plus que l'engorgement des services d'urgences hospitalières peut s'expliquer, en partie, par le manque d'implication des médecins libéraux dans la permanence des soins.

l'ordre et d'une équipe de médecins volontaires, mais aussi grâce à l'engagement de collectivités territoriales, qui participent à certains frais- locaux, vigiles, électricité. Seulement, aujourd'hui, ces médecins volontaires ont vieilli et ne trouvent pas de relève.

tenu de la détérioration de notre système de santé. En outre, ne croyez-vous pas qu'une généralisation du dispositif en 2022 est tardive ? Les urgentistes sont à bout !

que le rétablissement des gardes contribue à l'attractivité des territoires sous-dotés en praticiens libéraux. J'émets donc, à contrecoeur, un avis défavorable.

aux besoins actuels de la population. Toutefois, l'expression « en établissant des horaires de permanence des soins » introduit une forte ambiguïté sur le rôle dévolu aux SAS